La séance est ouverte.

Ces concours de lâches se propagent depuis plusieurs jours, relayés par les réseaux sociaux. La réponse à apporter doit être la fermeté. La nouvelle mode de ces criminels est de se filmer pendant leurs attaques contre les forces de l'ordre. Désoeuvrés ou protégeant des trafics, ils oublient bien vite la chance qu'ils ont de vivre dans un pays qui respecte l'État de droit et qu'eux-mêmes ont intérêt à respecter. Rien ne saurait justifier ces atteintes à l'ordre public, à la sécurité de nos concitoyens et à celle de ceux qui les protègent au quotidien les gendarmes, les policiers et les pompiers, à qui je veux rendre hommage. Les tensions dans les quartiers défavorisés sont en recrudescence. Voilà plus de trente ans que les gouvernements successifs tentent d'en venir à bout, sans y parvenir vraiment. Il semble qu'une trentaine d'individus était impliquée dans le guet-apens de Chanteloup-les-Vignes. Seules deux interpellations ont eu lieu à ce jour. Dans cette ville, comme ailleurs, cette situation n'est pas acceptable. La réponse judiciaire doit être à la hauteur des infractions commises. Monsieur le ministre de l'intérieur, je sais que vous vous êtes rendu sur les lieux hier matin. Que comptez-vous faire pour que les forces de l'ordre disposent de moyens plus importants, nécessaires à l'accomplissement de leur mission

La reconquête républicaine que nous devons conduire dans ces quartiers ne relève pas que de la seule police. Elle en relève, bien évidemment, mais elle relève aussi de l'ensemble de l'action portée sur ces territoires.

Chanteloup est une ville française comme Mantes, Béziers ou Brest, qui pansent leurs plaies et se battent au quotidien pour reconquérir, mètre carré par mètre carré, chaque morceau de leur territoire républicain que des criminels souhaitent voir disloqué. Lorsqu'on brûle nos villes, qu'on attaque nos policiers ou qu'on menace nos élus, c'est la République qu'on brûle, qu'on attaque et qu'on menace, monsieur le Premier ministre. Or, pour bien combattre ce mal, il faut bien le nommer et bien le comprendre. Relativiser ce qui s'est passé en qualifiant les agresseurs « d'imbéciles » fut une erreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces agresseurs, très organisés, défendent l'extraterritorialité de leur espace. Ils rejettent les lois de la République, ils refusent toute autorité venue de l'État, ils interdisent à la République de s'occuper de leurs affaires. Ils font scission, monsieur le Premier ministre. Sécession, plutôt ! C'est cela que vous devez nommer et combattre avec la plus grande fermeté.

La réponse est oui : j'ai la chance de connaître cette commune des Yvelines, ainsi que sa maire. Je m'y suis rendu en tant que Premier ministre. J'ai visité un certain nombre de quartiers, ainsi que le commissariat. J'ai pu rencontrer ceux qui, pour le compte des services de l'État et en tant qu'élus locaux,

Pour ce faire, nous essayons d'attaquer le problème de toutes les façons possible. Lorsque nous doublons le budget de l'ANRU, nous ne le faisons pas pour le plaisir de doubler un budget. Nous le faisons parce que, à l'écoute des élus locaux, nous savons que les opérations de rénovation urbaine sont des éléments puissants de réponse à ce problème. Je le sais, parce que j'écoute Mme la maire de Chanteloup-les-Vignes, parce que j'écoute, le cas échéant, le président du conseil départemental des Yvelines et parce que, madame la sénatrice, j'ai été maire du Havre

de façon théorique. Je sais que les opérations de rénovation urbaine permettent d'apporter non pas toutes, mais une partie des réponses que ces quartiers exigent. C'est exactement la même logique lorsque, avec l'ensemble du Gouvernement, nous essayons d'augmenter les effectifs de la police nationale

que l'éducation fonctionne mieux, y compris et surtout dans les zones dites sensibles, c'est exactement la même logique. Nous essayons d'aborder cette question par tous les bouts, si vous me permettez cette expression. Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté. Nous en avons discuté avec Mme la maire de Chanteloup-les-Vignes. Elle a d'ailleurs

nous venions perturber des trafics de stupéfiants à Chanteloup, comme dans d'autres villes. Lorsque l'on perturbe ces trafics, lorsque l'on vient

que nous allons poursuivre. La lutte contre le trafic de stupéfiants, la préparation du futur dans ces quartiers, dans ces villes, sont les objectifs du Gouvernement, et je suis sûr que vous les partagez.

Union Centriste. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État chargée des affaires européennes et concerne la visite du Président Emmanuel Macron en Chine. Le Président de la République a raison : seule l'Union européenne, dans une approche coordonnée, peut devenir « un partenaire crédible et efficace » de la Chine. la Chine. La France ne peut s'engager seule en Chine. Elle n'a pas la taille critique pour contrebalancer l'émergence de cette puissance aux aspirations dominatrices. S'il est légitime que la Chine veuille s'affirmer comme une grande puissance mondiale, elle trace son chemin largement à l'écart des règles du jeu occidentales, fondées sur la réciprocité des échanges, sur la transparence commerciale et sur la probité juridique. Ne parlons même pas de valeurs démocratiques ou de libertés publiques ... Le régime chinois construit un monde orwellien pour assurer l'unité de son peuple dans un espace clos par une « cybermuraille de Chine C'est au sein de ce monde hermétique que se développent leurs champions nationaux comme Huawei ou Alibaba. Il serait suicidaire pour l'Union européenne de continuer à laisser la Chine investir sur nos marchés sans bénéficier d'un principe de réciprocité. Ce qui est interdit à nos entreprises en Chine doit être interdit aux entreprises chinoises dans l'Union européenne. Comment pensez-vous imposer la réciprocité des échanges entre la Chine et l'Union européenne ?

fondées sur un respect mutuel de nos règles. La visite d'État du Président de la République en Chine qui s'achève aujourd'hui a permis de poursuivre et d'amplifier cette dynamique, impulsée également lors de la visite du Président Xi Jinping de Jean-Claude Juncker et d'Angela Merkel pour incarner cette dimension européenne et arriver à construire un partenariat eurochinois ambitieux, à la hauteur des différents enjeux, notamment, comme vous l'avez rappelé, en matière de protection des données personnelles.

pour la réplique. La Chine n'est pas un État de droit, mais un État de lois. Elle ne s'embarrasse pas de principes de transparence et de loyauté pour décrocher des marchés publics à l'international. Pour vendre en Chine, toute l'industrie cosmétique doit passer par le site Alibaba. On peut donc se demander quel sera l'avenir des brevets des molécules cosmétiques. Les entreprises européennes ont besoin de protection commerciale.

À la rentrée 2018, des évaluations en CP et CE1 ont été mises en place afin d'identifier les compétences acquises par les élèves, ainsi que leurs difficultés. En comparaison, les mêmes évaluations nationales réalisées cette année font apparaître, comme vous l'avez déclaré dimanche dernier, des « progrès significatifs » chez les enfants évalués progrès sur la fluidité de lecture et la capacité de calcul, progrès dans les territoires les plus défavorisés. Soyons clairs : dix des treize critères évalués en CE1 montrent une amélioration par rapport à l'année dernière, mais, en même temps, une faible majorité d'écoliers a acquis le niveau attendu en ce qui concerne la maîtrise des additions et des soustractions. Nous ne pouvons qu'espérer que ces progrès se confirmeront et s'amplifieront, et ce dans l'intérêt des enfants. Nous le souhaitons toutes et tous dans cet hémicycle. Aussi, afin que ces résultats s'inscrivent dans une dynamique positive sur le long terme, pourriez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur ce qui, selon vous, explique cette amélioration ?

Comme vous le savez, nous allons dédoubler les grandes sections de maternelle en REP et en REP+, de façon à ce qu'il y ait des classes de douze élèves, et améliorer le temps d'encadrement partout, en garantissant un maximum de vingt-quatre élèves par classe dans toute la France en grande section de maternelle, en CP et en CE1.

Il y a quelques jours, nous étions sur ces travées pour soutenir les élus, faciliter l'exercice quotidien de leur mandat et encourager leur vocation, au service de leurs concitoyens. Que souhaitent-ils ? Monsieur le ministre, vous me permettrez de citer votre collègue chargé des collectivités territoriales : « Si les élus souhaitent que nous corrigions les défauts des réformes passées, ils veulent aussi de la stabilité. » Je ne dirais pas mieux ! Toutefois, ce qui vaut en matière institutionnelle vaut aussi en matière de finances locales, car, pour assurer efficacement l'ensemble des services à la population, les communes et EPCI doivent disposer de réelles capacités d'action. En la matière, l'inquiétude est grande. En effet, élus et candidats, qui préparent leur programme municipal sur des bases crédibles, viennent de prendre connaissance des simulations des conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur le potentiel fiscal. Le mécanisme est pourtant bien connu : malgré une compensation à l'euro près, la suppression de la taxe d'habitation jouera nécessairement sur le potentiel fiscal et, donc, sur le niveau des dotations d'État et des péréquations correspondantes. Sont ainsi appelés à varier dès 2023, et donc en cours de mandat, près de onze des dix-huit critères de de répartition pour les communes. Nous sommes loin de la stabilité et de la visibilité fiscales nécessaires à l'exercice serein du mandat d'élu. Sur la base de ces simulations, les communes les plus pauvres deviendraient subitement plus riches, grâce à une hausse mécanique de leur potentiel fiscal, et donc moins aidées par l'État, tandis que des communes réputées plus riches, connaîtraient connaîtraient la trajectoire inverse ! Où est la logique fiscale ? Où est la solidarité nationale ? Où est l'esprit de la décentralisation ? Monsieur le ministre, mes interrogations sont donc simples : comment et quand comptez-vous concrètement corriger les effets néfastes des variations du potentiel fiscal ? Allez-vous accueillir les propositions des sénateurs, qui souhaitent rectifier dès maintenant les conséquences majeures induites par la fin de la taxe d'habitation ?

J'entends deux interrogations majeures : l'une sur la stabilité et la visibilité ; l'autre, plus technique, sur le potentiel fiscal servant de référence au calcul des critères d'accès à telle ou telle dotation. Sur la stabilité, nous pouvons rassurer les élus. Depuis le début de ce quinquennat, nous avons fait le choix de stabiliser les dotations à un niveau global : le budget pour 2020 prévoit la stabilité de la

Jacqueline Gourault et moi-même l'avons dit lors de notre audition par le Comité des finances locales, le 26 septembre dernier, et j'ai eu l'occasion de le redire voilà quelques jours devant la délégation aux collectivités territoriales de votre assemblée

que la suppression de la taxe d'habitation et la réforme de la fiscalité locale se traduisent par l'évolution artificielle d'un indicateur qui conditionne l'accès à telle ou telle dotation.

baisser de 20 % et 200 000 seront privés de toute indemnité ! Ce sont donc plus d'un million de personnes qui seront frappées de plein fouet. Croyez-vous sérieusement, madame la ministre, que cette demandeuse d'emploi qui a interpellé le Président Macron à La Réunion en lui disant « il n'y a pas de travail, comment fait-on avec 790 euros par mois ? »

pour ne prendre que quelques exemples. Votre réforme enfoncera la tête des plus précaires sous l'eau. C'est une réforme sexiste et anti-jeunes ! Les syndicats et les associations des personnes privées d'emploi sont vent debout contre cette réforme et appellent, très justement, à manifester le 30 novembre et le 5 décembre. Les agents de Pôle emploi se disent eux aussi choqués par ces nouvelles règles. Ma question est simple, madame la ministre. Avec cette réforme inique, vous comptez faire une économie de 4,5 milliards d'euros en trois ans. Pourquoi ne pas vous attaquer aux allégements de cotisations patronales, qui, de 2013 à 2019, ont atteint 26 milliards d'euros ?

Qu'est-ce que votre réforme ? C'est une machine à faire exploser la précarité et la pauvreté ! Plus de neuf millions de pauvres dans notre pays aujourd'hui, ne trouvez-vous pas que c'est suffisant ? N'est-ce pas inacceptable ? Pourquoi faire encore grossir leurs rangs ? Vous avez décidé de supprimer l'Observatoire national de la pauvreté. Madame la ministre, casser le thermomètre ne fait pas baisser la fièvre ! Votre politique

Pour ce gouvernement, le cap est clair : à droite toute ! Cette réforme, imposée par décret, est, pour reprendre les mots de Laurent Berger, « une des réformes les plus dures socialement qui s'est opérée ces vingt-cinq dernières années Avec les nouvelles conditions draconiennes d'accès aux droits, on estime que, en 2020, sur les 2,6 millions de personnes qui auraient bénéficié d'indemnités avec l'ancien système, près de 10 % ne pourront ouvrir aucun droit, et 23 % des bénéficiaires verront leurs droits rognés pour une question purement comptable. Eh oui ! Pis, au 1 avril 2020, avec votre nouveau mode de calcul, 1,4 million de demandeurs d'emploi verront leurs indemnités baisser drastiquement. Les personnes ayant un rythme de travail fractionné, déjà précaires, seront les premières impactées. Madame la ministre, vous faites des économies sur le dos des plus fragiles ! Vous culpabilisez les chômeurs, vous en faites des boucs émissaires, sans leur donner les moyens de retrouver un véritable emploi. Arrêtez cette politique de régression et de ségrégation ségrégation sociales ! Mettez en place des mesures ambitieuses pour résorber le chômage, lutter contre la précarité et accompagner réellement les chômeurs vers l'emploi

000 demandeurs d'emploi seront en formation. Nous investissons plus de 1 milliard d'euros dans l'insertion par l'économique dans le cadre du budget qui vous sera présenté dans quelques semaines. J'espère que vous le voterez, puisque, comme nous, vous souhaitez l'insertion des plus vulnérables. Nul n'est inemployable, mais il faut des marchepieds pour certains. En ce qui concerne

Si je parle avec de grands mots, madame la ministre, vous, vous parlez de façon technocratique et vous manquez singulièrement d'humanité. Derrière vos chiffres et vos statistiques, il y a des hommes et des femmes qui sont dans la misère sociale. Ce n'est pas en essayant de les monter les uns contre les autres ou en dénonçant l'assistanat que vous résoudrez

les cambriolages de 8 % et les violences sexuelles de 5 %. Pendant que la mairie de Paris et la préfecture de police se renvoient la balle, ce sont les Parisiens qui trinquent. Aucun territoire parisien n'est désormais épargné

Votre métier, ce n'est pas d'interpeller la société, c'est d'interpeller les délinquants. » Et je ne parle pas de la crise des « gilets jaunes » et des désagréments causés aux Parisiens

La lutte contre la délinquance n'est pas un sujet secondaire. En termes de doctrine sécuritaire, je ne connais que deux mots : la fermeté et le résultat.

d'ordre public, de patrouiller comme des effectifs de sécurité publique, quand ils n'ont pas de missions d'ordre public à accomplir. Il s'agit d'une réforme importante, qui se traduit par des effectifs supplémentaires sur la voie publique. Ce n'est pas vrai ! Par ailleurs, nous souhaitons un meilleur équilibre dans la répartition des tâches entre ce qui relève de la préfecture de police en matière d'encadrement de manifestations récréatives, sportives ou culturelles et ce qui doit relever de la Ville de Paris. Ce travail est en cours, mené par le préfet de police. Le deuxième pilier est constitué par les investigations judiciaires.

Madame la ministre, j'ai eu l'occasion de vous alerter sur les difficultés rencontrées par les transporteurs de passagers et de marchandises sur nos routes. Ils ne peuvent exercer pleinement leur métier.

: une véritable indépendance du Liban et l'établissement d'un État laïque. La France est depuis longtemps un pays ami du Liban. Comment Comment comptez-vous répondre aux attentes du peuple libanais, qui aspire à un système politique moins corrompu et à une amélioration de la situation économique ?

nous ne sommes pas dans l'ingérence, mais nous suivons avec la plus grande attention la situation au Liban, marquée par d'importantes manifestations de citoyens réclamant quotidiennement, depuis plusieurs semaines, des réformes sur les plans économique, social et politique.

et les manifestations qui ont conduit à la démission du Premier ministre Saad Hariri, le 29 octobre, montrent que la suite est incertaine et que c'est d'abord aux Libanais de l'écrire. La France insiste sur l'importance de la stabilité du pays dans un contexte régional très tendu, d'une part, et appelle à écouter les manifestants et à leur répondre, d'autre part, leur demande de réformes nous semblant légitime. À la suite de la démission du Premier ministre, il nous paraît essentiel qu'un gouvernement puisse rapidement être formé pour conduire les réformes dont le pays a besoin. Dans le contexte de crise économique, sociale et politique que connaît le Liban, il revient aux responsables politiques libanais de faire prévaloir un esprit d'unité nationale et de responsabilité pour garantir la stabilité, la sécurité et l'intérêt général du pays. Dans cet esprit, tout doit être fait pour éviter les provocations et les violences, ainsi que pour préserver le droit des citoyens à manifester pacifiquement. Il est donc essentiel que l'ensemble des forces politiques facilitent dès à présent la formation d'un nouveau gouvernement qui puisse répondre aux aspirations légitimes exprimées par les Libanaises et les Libanais et prendre les décisions indispensables au rétablissement économique du pays. La France, dans le cadre fixé par la conférence CEDRE, se tient prête à soutenir le Liban. Dans ce moment crucial, la France, comme toujours, se tient aux côtés du peuple libanais.

Madame la ministre, nous approuvons l'objectif de libérer du temps médical pour faciliter l'accès aux soins. Cette politique publique implique, d'une certaine manière, un partage des compétences entre professionnels. les infirmiers peuvent être formés aux pratiques avancées et les pharmaciens peuvent désormais contribuer aux campagnes de vaccination antigrippale, mais ce nouveau partage des compétences, que nous appelons de nos voeux, est source d'incompréhension et, parfois, d'un sentiment d'inégalité.

formellement, l'acte de vaccination antigrippale est facturé de la même manière, qu'il soit effectué par un pharmacien ou par un infirmier, force est de constater que la rémunération de 6,30 euros n'est effective

La France s'est dotée d'une stratégie globale en matière de lutte contre la grippe, pour protéger par tous les moyens les publics vulnérables, éviter des hospitalisations, des décès, et préserver nos services des urgences. Après avis de la Haute Autorité de santé, j'ai souhaité harmoniser les compétences des professionnels de santé impliqués dans la vaccination contre la grippe, que ce soit les sages-femmes, les infirmiers ou les pharmaciens. Nous avons autorisé la vaccination par les pharmaciens dans deux régions en 2017, puis dans quatre régions en 2018. Au regard des résultats des évaluations et des bénéfices pour la santé publique, j'ai décidé de généraliser à toute la France le dispositif pour cette campagne vaccinale. S'agissant S'agissant des infirmiers, alors qu'ils ne pouvaient pas réaliser la primo-vaccination, j'ai supprimé cette limitation depuis la campagne hivernale 2018-2019.

Dans le même temps, les infirmiers libéraux peuvent également facturer les indemnités de déplacement si les actes de vaccination sont pratiqués à domicile. La politique de prévention et de santé que je mène englobe

Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le ministre, le public présent dans cet hémicycle ne peut ni applaudir ni conspuer les orateurs. La raison en est simple : les élus ne légifèrent pas sous la menace C'est un principe essentiel dans une démocratie. Depuis le vote, par notre assemblée, d'une proposition de loi visant à interdire le port de signes religieux lors des sorties scolaires,

est jetée en pâture. Un groupe Facebook parle même de « sénateurs nazis » et invite ses membres à communiquer les lieux de résidence et les photos des parlementaires qui ont voté ce texte ... Les intimidations sont explicites.

a été contrainte, devant la violence des attaques, de se constituer partie civile. Je tiens lui apporter tout mon soutien. Un texte a été démocratiquement voté par une assemblée, des parlementaires sont traqués, menacés, mais, monsieur le ministre, on ne vous a pas entendu on ne vous a pas entendu dénoncer ce qui constitue une atteinte grave à l'exercice d'une démocratie sereine. Pourquoi ce silence ? Veuillez Vous êtes le ministre de l'intérieur. À ce titre, quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à ces tentatives d'intimidation ? Devons-nous nous inquiéter ? La parole

Au 1 septembre, nous avions enregistré 244 actes de violence ou de malveillance à l'égard d'élus ou de parlementaires : 212 dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes » et 32 dans celui de la

Au nom du groupe RDSE, je souhaite saluer l'excellent travail accompli par nos collègues Laurent Lafon et Jean-Yves Roux dans le cadre de la mission d'information sénatoriale sur les nouveaux territoires de l'éducation.

de pratique culturelle ou sportive. Je parle ici de 36 % de nos écoles et de 20 % de nos élèves. La réalité d'aujourd'hui et les projections démographiques pour demain démontrent que l'offre scolaire de proximité dans ces territoires ruraux est un sujet à traiter prioritairement. Je vous propose donc de ne pas attendre, monsieur le ministre, pour faire évaluer les propositions de nos collègues, dans la perspective de leur application. Évaluer l'indice d'éloignement géographique permettrait de mieux valoriser le travail des enseignants dans ces territoires et de rendre plus attractifs des postes aujourd'hui délaissés. En Gironde, le dialogue de confiance qui s'est instauré entre les collectivités locales et l'éducation nationale déconcentrée s'est révélé décisif pour construire une offre scolaire adaptée aux réalités du terrain.

socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Le 31 août dernier, à Villeurbanne, un jeune homme a été tué par un migrant afghan aux motivations mêlant délire religieux et troubles psychiatriques graves. Ce drame atroce illustre la nécessité de soins psychiatriques adaptés pour tous, y compris les migrants. Or aujourd'hui, vous annoncez des mesures visant à durcir les conditions d'accueil

D'abord, un risque sanitaire : nous parlons de personnes qui souffrent parfois de maladies infectieuses. Faut-il attendre que leurs pathologies s'aggravent pour les prendre en charge ? En durcissant l'accès aux soins, ne faites-vous pas peser un risque sanitaire sur tous ? Ensuite, un risque juridique : la France a ratifié la directive Accueil de l'Union européenne, dont l'article 19 précise que les États membres doivent assurer les soins médicaux urgents et le traitement des maladies psychiatriques des demandeurs d'asile. Monsieur le Premier ministre, cette mesure est-elle conforme aux engagements européens de la France ?

la ministre, lutter contre tous les abus, qui peut y être opposé ? Mais, en l'occurrence, vous prenez des mesures envers les plus démunis qui pénalisent l'ensemble des migrants et nous font prendre un risque sanitaire. En matière de santé, il faut rester simple : mieux

Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme la ministre des armées. À la veille des cérémonies mémorielles du 11 novembre, les représentants du monde combattant sont en émoi En effet, le devenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) est plus qu'incertain. Alors même que le champ d'intervention de l'ONAC-VG s'est considérablement étendu, notamment avec la prise en compte des victimes du terrorisme, le projet de budget pour 2020 prévoit de lourds transferts de charges vers sa trésorerie. En l'état actuel de la réorganisation de l'ONAC-VG, la débudgétisation ainsi opérée n'est pas soutenable. Au moment où la restauration de l'unité nationale devrait être une urgence, au moment où le souvenir de nos glorieux aînés devrait être un exemple, vous laissez Bercy étouffer leur mémoire ! Que comptez-vous faire, madame la ministre, pour enrayer cette dangereuse évolution ?

et de solidarité pour le monde combattant, ainsi que notre opérateur principal en matière d'action mémorielle sur les territoires. Vous avez évoqué les mesures inscrites dans le projet de loi de finances pour 2020 et les craintes qu'elles peuvent susciter. Je veux aujourd'hui vous rassurer pleinement à cet égard. Les mesures d'économie prévues, pour un montant de 2 millions d'euros, qui comportent des réductions d'effectifs, sont liées à la mise en place d'une dématérialisation, à la baisse du nombre de bénéficiaires et à la réorganisation des fonctions de l'administration centrale. Cette évolution, je vous le rappelle, a été votée par le conseil d'administration de l'ONAC-VG, représentants des organisations syndicales. Il n'y a pas eu d'opposition parce qu'elle n'affecte pas le réseau départemental de l'office, qui sera maintenu dans son intégralité, les fonctions d'accueil étant évidemment préservées.

Vous l'aurez compris, le Gouvernement est particulièrement attentif à la préservation de l'ONAC-VG, dont les missions sont indispensables, qu'il s'agisse de l'accompagnement des anciens combattants et des victimes d'attentats dans notre pays ou de la préservation de la mémoire combattante. La parole je convoque la mémoire et vous invoquez la comptabilité ! Sauf votre respect, cette réponse n'est pas au niveau. Alors que le brigadier-chef Ronan Pointeau a trouvé la mort en opération au Mali à l'âge de 24 ans, samedi dernier,

la séance. Elle sera reprise à dix-sept heures quinze, à l'issue de la conférence des présidents, pour l'examen de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. La séance est suspendue.

La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance. Par ailleurs, je vous informe que le Gouvernement

que son groupe entendait déposer prochainement une proposition de loi sur les violences à l'intérieur de la famille, soit exactement le même sujet

de la protection contre les violences au sein du couple. Vous le savez, cette proposition de loi porte sur deux thématiques essentielles : les ordonnances de protection, dont nous voulons accélérer le traitement,

le Grenelle des violences conjugales, qui a été lancé le 3 septembre dernier par le Premier ministre et qui sera clôturé le 25 novembre prochain,

aujourd'hui soumise. C'est encore dans cet esprit que nous souhaitons aborder les débats qui vont se tenir dans cet hémicycle, afin que soient

Dans la lutte contre les violences conjugales, la justice occupe évidemment une position centrale. Je mène à ce titre, depuis plusieurs mois, une politique extrêmement volontariste, construite autour d'un plan d'action très structuré. Ma circulaire du 9 mai dernier ainsi rappelé aux procureurs le caractère prioritaire du traitement de ces violences, en les incitant à utiliser pleinement l'arsenal législatif dont ils disposent, comme les téléphones grave danger (TGD) ou l'ordonnance de protection, des dispositifs qui méritent d'être mis en lumière. Je souhaite bien entendu que le recours au dispositif de l'ordonnance de protection soit facilité, afin que sa mise en oeuvre devienne une pratique très régulière, dès que la situation dont le juge est saisi correspond au cadre pour lequel elle est prévue. Mes services ont d'ailleurs analysé toutes les décisions d'ordonnance de protection qui ont été rendues depuis 2016, soit au total 3 102. Ce chiffre est d'ailleurs très inférieur au nombre d'ordonnances de protection délivrées en Espagne.

Un guide très complet exposant l'objectif et le cadre juridique de cette mesure a été réalisé par la direction des affaires civiles et du sceau de mon ministère. Il sera très rapidement et très largement diffusé. La mise en place du bracelet anti-rapprochement (BAR) pour les auteurs de violences conjugales à titre de peine, mais aussi avant tout jugement pénal dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ou hors de toute plainte dans le cadre civil d'une procédure d'ordonnance de protection, a été annoncée par le Premier ministre dès l'ouverture du Grenelle. Cette mesure fait l'objet d'un très large consensus. J'avais moi-même d'ailleurs engagé des travaux en ce sens avec plusieurs parlementaires- je pense notamment aux députés Guillaume Vuilletet, Guillaume Gouffier-Cha et Fiona Lazaar. Le groupe LaREM de l'Assemblée nationale avait également déposé une proposition de loi qui traduisait ce travail. Je suis ravie que, dans un esprit de coconstruction, il ait finalement été décidé, pour avancer plus rapidement, d'opter pour l'examen de la proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Parce que le phénomène des violences au sein du couple est très spécifique, parce que certains mécanismes psychologiques, tels que l'emprise, n'ont été clairement identifiés et décrits que depuis quelques années, j'ai souhaité renforcer l'offre de formation en la matière. Un important travail a donc été réalisé en ce sens, et l'École nationale de la magistrature offre, depuis le début de ce mois, de nouvelles formations ouvertes aux magistrats, mais aussi aux personnels de l'administration pénitentiaire ou encore de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'à des officiers de police judiciaire, à des avocats et à des personnels associatifs, sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est que les magistrats soient parfaitement formés et sensibilisés au traitement spécifique de cette délinquance. tous les magistrats qui seront amenés à changer de fonction devront suivre un module de formation sur les violences conjugales -j'y insiste, cette formation sera obligatoire. Au-delà de ces questions, il me paraît essentiel de travailler au développement d'une meilleure synergie entre tous les acteurs. J'ai eu l'occasion de le dire, il faut

C'est pourquoi une expérimentation a été lancée au tribunal de grande instance de Créteil, juridiction pilote, aux fins d'élaborer un schéma modèle de traitement judiciaire des faits de violences conjugales, intégrant tout à la fois l'urgence des réponses et la prise en considération de leur particularité. Deux autres juridictions, de taille plus réduite, deviendront, elles aussi, pilotes en la matière, afin que le système retenu soit applicable à l'ensemble des tribunaux

C'est dans cet esprit que j'ai installé, à la Chancellerie, un groupe de travail réunissant l'ensemble des acteurs concernés. Ce groupe suivra, au-delà même du Grenelle, l'avancée des actions annoncées.

en réponse à M. Jean-Pierre Sueur. Pour en revenir plus précisément aux dispositions de la proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui, je rappelle que ce texte vise, d'une part, à renforcer l'ordonnance de protection,

inciter non seulement les parties, mais encore les avocats qui les assistent, à demander les mesures prévues par les textes, ainsi qu'à renforcer ces mesures.

Pour cette raison, le rappel du principe selon lequel la délivrance d'une ordonnance de protection n'est pas subordonnée à une plainte préalable a une vertu pédagogique. Le texte qui vous est présenté conforte aussi le traitement de l'urgence. L'Assemblée nationale a en effet adopté un amendement visant à instaurer « un délai maximal de six jours à à compter de la fixation de la date de l'audience » pour que le juge aux affaires familiales rende sa décision. Je crois qu'il est effectivement indispensable de raccourcir les délais de délivrance des ordonnances de protection. Il est toutefois tout aussi nécessaire de respecter le principe du contradictoire et la nature spécifique de la procédure civile, qui repose, je le précisais à l'instant, sur la volonté des parties, donc sur des principes différents de ceux du procès pénal.

Par ailleurs, ainsi que je m'y étais engagée dès le mois de mai dernier, le juge aux affaires familiales pourra prononcer la pose d'un bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l'ordonnance de protection. Le Gouvernement a travaillé de concert avec les parlementaires pour sécuriser ce dispositif, ordonné dans un cadre civil, l'accord du défendeur étant requis pour éviter tout risque constitutionnel. À défaut d'accord de sa part, le dossier sera transféré au procureur de la République, qui pourra mettre en oeuvre les poursuites pénales. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je me félicite de ce dialogue parlementaire constructif. Je suis certaine que la loi qui en sera issue contribuera à assurer une meilleure protection des victimes de violences au sein de la famille. En ce sens, il me tient particulièrement à coeur que ce dispositif soit opérationnel dans les meilleurs délais.

De très nombreux contributeurs et des groupes de travail réfléchissent actuellement aux moyens de renforcer encore la protection des victimes de violences. Bien évidemment, je suis

En conclusion, je tiens à vous assurer que l'engagement du ministère de la justice est absolu et que nous continuerons, avec l'aide de tous- non seulement les forces de l'ordre, mais aussi les avocats, les réseaux associatifs et l'ensemble de la société civile -, à lutter contre ces actes qui, en meurtrissant chaque jour

De nombreux drames pourraient être évités si une action efficace était conduite par les pouvoirs publics dès le signalement des premiers faits de violence. Le 3 septembre dernier, le Gouvernement a lancé un Grenelle des violences conjugales, qui se prolongera jusqu'au 25 novembre prochain, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Sans attendre les conclusions du Grenelle, le Gouvernement a rendu publiques une dizaine de mesures d'urgence. elles nécessite une intervention du législateur, ce qui explique que nous soyons saisis de cette proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. Déposée par notre collègue député Aurélien Pradié, qui en a également été le rapporteur, cette proposition de loi a été adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale, le 15 octobre dernier. de ce vote, l'Assemblée nationale a montré que la représentation nationale pouvait se rassembler, par-delà les clivages partisans, autour de cette grande cause qu'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Sur ce sujet, certains États ont été précurseurs, notamment l'Espagne, qui s'est dotée, voilà une dizaine d'années, de juridictions spécialisées et d'un dispositif anti-rapprochement qui a fait ses preuves. L'introduction en France du bracelet anti-rapprochement constitue la mesure phare de cette proposition de loi. Le texte propose d'autoriser son utilisation à toutes les étapes de la procédure pénale au moment de la condamnation, notamment dans le cadre d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, à l'occasion d'une mesure d'aménagement de peine, par exemple une libération conditionnelle, mais aussi pendant l'enquête, lorsque la personne mise en cause est placée sous contrôle judiciaire. Chaque fois, ce sera un magistrat du siège qui prendra la décision d'ordonner le recours au bracelet anti-rapprochement. Ce bracelet, attaché à la cheville du conjoint violent, et le boîtier, confié à la victime, permettent de géolocaliser en permanence l'un et l'autre, et de déclencher une alerte dans un centre de surveillance s'ils s'approchent trop l'un de l'autre. Il s'agit donc d'un outil de prévention, destiné à éviter la répétition des violences. Pour favoriser le recours à ce dispositif, il est prévu d'informer les victimes, au moment du dépôt de plainte, qu'elles pourront en bénéficier. En théorie, le conjoint violent pourra refuser de porter ce bracelet, mais son refus pourra entraîner la révocation, par le juge, de la mesure dont il bénéficie, et donc son incarcération ou son placement en détention provisoire.

Nous ne pouvons toutefois que regretter que les deux expérimentations votées par le législateur, en 2010 et en 2017, n'aient jamais été suivies d'effet, alors que certaines juridictions- je pense en particulier au tribunal de Pontoise -étaient prêtes à les mettre en oeuvre.

par tout moyen » ; ensuite, elle introduit un nouveau cas dans lequel l'attribution du TGD serait autorisée, en cas d'urgence. La proposition de loi comporte ensuite un volet de droit civil, qui vise essentiellement à améliorer le dispositif de l'ordonnance de protection, introduite dans notre législation en 2010. L'ordonnance de protection est délivrée, en urgence, par le juge aux affaires familiales, lorsque celui-ci estime vraisemblable que des faits de violence aient été commis au sein du couple et s'il pense que la victime ou un ou plusieurs enfants restent exposés à un danger. Dans le cadre de l'ordonnance de protection, le juge peut prendre des mesures civiles assez classiques, par exemple en matière d'autorité parentale ou de résidence séparée. Il peut aussi prendre des mesures de protection de la victime, par exemple pour la faire bénéficier, sans délai, de l'aide juridictionnelle. Il peut enfin décider de mesures à connotation pénale, imposées à l'auteur des violences, exemple l'interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes ou encore l'interdiction de détenir ou de porter une arme. Pourtant, le nombre demandes d'ordonnance de protection reste faible

Dans ce contexte, la proposition de loi cherche à lever les obstacles à la délivrance de ces ordonnances, en rappelant notamment que le dépôt d'une plainte ne peut être exigé. Dans le dessein d'accélérer leur délivrance, le texte prévoit également de fixer au juge l'ordonnance devrait être rendue dans les six jours qui suivent la fixation de la date de l'audience. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur cette question du délai au cours de l'examen des amendements. Enfin, le texte donne de nouvelles prérogatives au juge aux affaires familiales : ce magistrat pourrait interdire au conjoint violent de paraître en certains lieux et ordonner, à condition que les deux parties l'acceptent, le port d'un bracelet électronique anti-rapprochement. Ces dispositions créatives accentuent le caractère hybride de l'ordonnance de protection, à mi-chemin entre le droit civil et le droit pénal. Il n'est pas certain que les

Toutefois, la commission n'a pas voulu faire obstacle à l'entrée en vigueur de ces dispositions, qui renforcent malgré tout la position des conjoints victimes. Elle a seulement souhaité donner un caractère temporaire à l'utilisation du bracelet anti-rapprochement en matière civile, qu'elle juge particulièrement innovante au bout de trois ans, sur le fondement d'une évaluation, nous pourrons prolonger cette mesure ou la faire évoluer si les doutes exprimés se révélaient fondés. J'en terminerai en évoquant les mesures destinées à faciliter le relogement des femmes victimes de violences conjugales. Vous le savez, la loi fait de l'éviction du mari violent du domicile conjugal la règle de principe. Il peut arriver néanmoins que la victime ne souhaite pas regagner son domicile, soit parce qu'il est associé à des souvenirs traumatiques, soit parce qu'elle juge plus prudent de déménager. Pour l'essentiel, le texte prévoit de mener, pendant une durée de trois ans, deux expérimentations. La première consiste à mettre en place un mécanisme de sous-location temporaire de logements relevant du parc social : des associations d'aide aux victimes se verraient confier la gestion de logements sociaux, qu'elles pourraient sous-louer, sous condition de ressources, aux femmes qui s'adressent à elles. La seconde vise à créer un dispositif d'accompagnement adapté en s'appuyant sur des mécanismes existants, comme la garantie locative Visale, qui permet de couvrir des impayés de loyers, ou le Loca-Pass, qui permet de financer le dépôt de garantie. Vous le voyez, mes chers collègues, ce texte apporte des réponses concrètes aux difficultés que rencontrent les femmes victimes de violences conjugales.

Je ne doute pas que le Gouvernement saura mobiliser les moyens budgétaires nécessaires pour assurer la réussite de ces nouvelles mesures. Il est possible que nous ayons à débattre à nouveau, au cours des prochains mois, de la question des violences faites aux femmes, car le Grenelle des violences conjugales devrait faire émerger d'autres propositions relevant du domaine législatif. Vous pourrez toujours compter sur nous, madame la garde des sceaux, pour les examiner avec sérieux, en veillant chaque fois à concilier le nécessaire volontarisme dans la lutte contre les violences faites aux femmes avec le souci de l'efficacité et de la préservation des principes fondamentaux qui garantissent notre liberté à tous.

le 3 juillet dernier, plus de 150 sénateurs et sénatrices de tous les groupes publiaient dans un grand quotidien national, sur l'initiative de la délégation aux droits des femmes, une tribune sur les féminicides- un mot terrible qu'une actualité révoltante a, jour après jour, fait entrer dans notre vocabulaire. Ces femmes tuées ne sont pas des statistiques », écrivions-nous. « Elles ont des visages, des prénoms. Derrière les chiffres, il y a des enfants qui grandiront sans leur mère, des parents qui vieilliront sans leur fille. » Les victimes étaient alors au nombre de 71 depuis le

dit, on peut aussi déplorer que cette volonté politique ait tant tardé à s'exprimer, alors que la sonnette d'alarme était tirée depuis très longtemps par les experts et les acteurs de terrain. Prêter attention plus tôt à ces alertes aurait évité la mort à des centaines de femmes et aurait changé le destin de centaines d'enfants. On peut aussi s'interroger sur un calendrier qui empêche la prise en compte, par la future loi, des enseignements qui ne manqueront pas d'émerger du Grenelle des violences conjugales, dont la fin est prévue dans trois semaines environ. Ne devrons-nous pas, à la suite du Grenelle, débattre d'un nouveau texte législatif, alors que l'encre de la loi dont nous discutons aujourd'hui sera à peine sèche ? En dépit de cette réserve, relative à la méthode et non au fond, permettez à la délégation aux droits des femmes de se féliciter, par ma voix, que la proposition de loi traduise des recommandations recommandations que nous formulons régulièrement dans nos travaux sur les violences au sein des couples. Je pense notamment à la nécessité de proscrire toute tentative de médiation par le juge aux affaires familiales, dès lors que des violences ont été alléguées- et non commises -par l'un des parents. Très bien ! Quant au bracelet anti-rapprochement, il s'agit certainement d'un outil prometteur pour empêcher le passage à l'acte de l'auteur de violences. Gardons-nous toutefois de le considérer comme une « baguette magique » qui, à elle seule, mettrait fin au fléau des violences conjugales. Il est heureux que la commission des lois souhaite mettre à l'épreuve cet outil, qui sera aux mains du juge civil. Le suivi de cette mesure sera donc essentiel, et les moyens qui seront attribués à sa mise en oeuvre devront être à la hauteur des enjeux. En tant que parlementaires, nous devrons exercer notre vigilance lors du contrôle de l'application de la future loi. En matière de violences, l'outil répressif ne suffit pas, c'est une évidence. La prévention est essentielle, comme la délégation aux droits des femmes ne manque jamais de le souligner. Les meilleures lois, les outils les plus performants ne sauraient être efficaces si le personnel appelé à les appliquer et à les utiliser- policiers, gendarmes, magistrats -n'est pas formé à la psychologie des victimes et à l'emprise qu'exerce l'auteur des violences sur sa famille. En outre, l'effort de formation aux violences, qui est réel et mobilise beaucoup d'énergies- il convient d'en saluer les acteurs -, ne sert à rien

Leurs subventions sont désormais calculées au plus juste. Les bracelets électroniques et les téléphones grave danger seront inutiles si les associations ne peuvent plus accueillir, conseiller et orienter

À ces points de vigilance s'ajoute la nécessité de prêter une attention spécifique aux violences subies par les femmes handicapées ; c'est encore un sujet tabou. Veillons à ne pas faire de ces victimes particulièrement vulnérables les oubliées de la dynamique qui s'engage actuellement contre les violences. Enfin, les violences intrafamiliales imposent de réfléchir au maintien de l'autorité parentale, car un mari violent ne saurait être un bon père et un enfant témoin est toujours un enfant victime. victime. N'ayons pas la naïveté ou la suffisance de croire que l'adoption de cette loi nous dédouanera de nos responsabilités à l'égard d'un fléau qui touche tant de familles. C'est à une mobilisation de la société tout entière, dans tous les territoires et dans la durée, que nous appelle le glaçant décompte des féminicides. C'est notre responsabilité d'élus, de parents et de citoyens. En dépit de ces quelques interrogations et réserves, la délégation salue un texte qui marquera, nous l'espérons, une étape positive pour agir concrètement contre les violences conjugales.

de vies anéanties. Ce chiffre est insensé, insupportable ; il cache des douleurs insondables. Pourtant, il ne fait qu'approcher la réalité sans vraiment en rendre compte. Combien de femmes souffrent à l'heure où je m'exprime devant vous ? Combien sont gravement blessées ? Combien se sont suicidées ? 129 femmes tuées signe l'échec de toute une société, notre échec collectif. Devant ce drame quotidien, agir résolument contre les violences et les féminicides est une obligation. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale qui tend à agir contre ces violences, bien souvent constatées dans le cadre privé du foyer. Son adoption à l'unanimité montre montre que l'ensemble des députés, quelle que soit leur sensibilité, sont convaincus de la nécessité d'agir pour enrayer ce fléau. Pourtant, la situation dans laquelle nous nous trouvons cet après-midi ne doit pas manquer de nous interpeller. C'est bien une proposition de loi que nous examinons. Pour un sujet présenté il y a deux ans et demi comme la « grande cause du quinquennat », le recours à ce véhicule législatif a en soi une signification.

Je le dis donc sans détour : les conditions ne sont pas réunies pour garantir aux Françaises et aux Français une production qualitative de la loi ; je le déplore. Compte tenu des enjeux, puisqu'il s'agit bien d'épargner des vies, nous ne saurions nous en satisfaire. Je le disais à cette tribune en juillet 2018, à propos du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la « grande cause du quinquennat » débouche parfois sur de bien petites lois. Je crains que cela ne soit encore le cas aujourd'hui, alors qu'un tel sujet mérite, au contraire, un vaste projet de loi, impliquant les services de police et de gendarmerie, les services sociaux, les collectivités locales, la formation des agents et l'organisation judiciaire, en particulier la répartition des compétences entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des libertés et de la détention. Enfin, un projet de loi à la hauteur des ambitions affichées par le Président de la République lui-même exigerait que des moyens financiers massifs soient déployés afin d'améliorer la prise en charge des victimes, le soutien aux associations, l'hébergement d'urgence des victimes, la formation des personnels

de la possibilité d'ordonner le port de celui-ci en phase pré-sentencielle, bien qu'il s'agisse d'une mesure attentatoire aux libertés et que le texte fasse reposer cette décision sur le juge aux affaires familiales. C'est aussi le sens des mesures d'aide au logement, qui tendent à préserver de la précarité les victimes et, bien souvent, leurs enfants.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous commençons aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, un objectif qui, bien qu'il soit aujourd'hui consensuel,

Comment expliquer les réticences institutionnelles à sanctionner des actes connus de tous et décrits parfois crument dans la littérature ? Qui n'a appris, à l'école, le zeugma : « il battait la campagne et sa femme

à plus de 99 000 exemplaires en 1902 : « Alors, ce fut abominable. Cet aveu qu'il exigeait si violemment venait de l'atteindre en pleine figure, comme une chose impossible, monstrueuse. [ ...] Il la jeta d'une secousse en travers du lit,

à savoir la réticence à s'immiscer judiciairement dans la cellule conjugale au motif d'en préserver l'équilibre. Au contraire, l'immunité familiale s'est parfois renforcée après la publication de, avec la pénalisation de l'adultère ou de l'avortement et la reconnaissance d'un « devoir conjugal », c'est-à-dire la légalisation du viol entre époux.

dotions de nouveaux moyens techniques, avec le port d'un bracelet anti-rapprochement par les personnes condamnées. Enfin, il tend à faciliter la mise en oeuvre pratique de l'éloignement de la victime et son accès à un logement. La plupart de ces dispositions nous semblent aller dans le bon sens, de même que les modifications apportées par la commission des lois après les travaux importants réalisés par Mme la rapporteur, que je félicite et remercie. malgré sa vigilance, nous ne sommes pas convaincus de la pertinence du développement du recours au bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l'ordonnance de protection, surtout à titre expérimental, compte tenu des restrictions budgétaires que connaît le ministère de la justice. nous nous inquiétons qu'une telle mesure coercitive, prise par un juge civil en amont de toute condamnation, se heurte aux fondements de notre droit pénal. L'ordonnance de protection ne doit pas se substituer au procès pénal. C'est pourtant le chemin que nous prenons, sans doute en raison du manque de réactivité de nos juridictions, lié à leur manque de moyens. Nous proposons, au contraire, d'élargir les éléments fondant la prise d'une ordonnance de protection, afin que le doute profite toujours aux personnes dénonçant des violences, mais de limiter, dans le même temps, les conséquences coercitives pour les présumés auteurs de violences, qui devraient intervenir après le procès pénal seulement. Une demande d'ordonnance de protection sur deux échoue aujourd'hui faute de preuves suffisantes.

Tous ces facteurs altèrent la qualité de la communication au sein de la cellule familiale. À côté des solutions développées pour les victimes, des dispositifs d'écoute devraient également être mis en place en amont pour les personnes traversant ces difficultés, afin de prévenir tout basculement vers la violence. La dimension territoriale ne devrait pas être oubliée : c'est parfois un facteur aggravant, quand la ruralité accroît l'isolement. Des solutions innovantes ont d'ailleurs été développées sur le terrain, avec le financement de bus d'aide aux victimes. Du point de vue des capacités d'hébergement, les îles intérieures de la République pourraient utilement servir de refuges accueillants Enfin, et surtout, vouloir combattre la violence au sein de la famille sans évoquer celle qui s'exerce sur les enfants, qu'ils soient témoins ou victimes, me paraît un contresens énorme. On le sait, une part importante de ces enfants deviendront malheureusement des auteurs ou des victimes de violences familiales. Un récent rapport, produit par trois inspections générales, a justement formulé des propositions destinées à renforcer la lutte contre les morts violentes d'enfants. Nous proposerons des amendements qui s'en inspirent.

En conclusion, l'intolérance à l'égard des violences doit infuser à tous les niveaux de la société française, et la libération de la parole doit aboutir à des décisions de justice conformes aux grands principes de notre État de droit.

129 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint ! Autant de drames, avec des conséquences inimaginables pour les enfants et les familles. Autant de catastrophes, qui appellent des réponses concrètes et renforcées, des réponses qui s'appliquent vite- le plus tôt possible, afin d'éviter le pire -, des réponses qui prennent en compte les situations sociales et territoriales diverses des victimes, des réponses qui éloignent, qui protègent et qui donnent le temps de la reconstruction, des réponses efficaces au quotidien, qui enrayent la spirale infernale de la violence aveugle. Ces dernières années, des décisions ont été prises. Elles étaient bienvenues. Il faut maintenant, collectivement, aller plus loin. Depuis 2017, le Gouvernement a pris des initiatives politiques en la matière. Je pense à la mise en place du numéro d'appel 3919, Violences Femmes Information. Nous devons toutes et tous faire connaître au maximum ce numéro national de référence, mis en place afin d'écouter, d'informer et d'orienter des victimes vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. En conclusion du Grenelle ouvert en septembre dernier, les groupes de travail constitués dans ce cadre propositions destinées à lutter contre les violences faites aux femmes. Des mesures d'urgence ont d'ores et déjà été annoncées. Certaines relèvent de la compétence réglementaire, comme l'ouverture de 1 000 nouvelles places d'hébergement, l'audit des commissariats et des gendarmeries pour évaluer les conditions d'accueil ou encore l'ouverture de la possibilité de déposer plainte dans les hôpitaux. Ma collègue la députée girondine Bérangère Couillard, qui a copiloté les « grenelles locaux », évoquait hier, dans, l'exemple de la la cellule d'accueil d'urgences des victimes d'agression (Cauva) mise en place au sein du CHU de Bordeaux. Elle a par ailleurs remis ses conclusions hier. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre prochain, seront annoncées, au regard de ces importants travaux de consultation, de nouvelles mesures et de nouvelles actions. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ce cadre.

réduire les délais de délivrance des ordonnances de protection et à rendre ainsi ces dernières plus efficaces. Elle prévoit d'élargir le port du bracelet anti-rapprochement de l'auteur de violences dans le cadre du couple. Ce système permettra de géolocaliser et de maintenir à distance les conjoints ou ex-conjoints violents par le déclenchement d'un signal, selon un périmètre d'éloignement fixé par un juge.

renforcer l'hébergement d'urgence, en faisant du maintien de la victime dans le logement familial et de l'éloignement de l'auteur des violences la règle. Il renforcera l'outil que constitue le téléphone grave danger,

parentale lorsque l'un des deux parents est décédé des suites d'un homicide volontaire et que les faits mettent en cause l'autre parent, cela dès la phase d'enquête ou d'instruction

Elle nous a permis de participer à de nombreuses auditions très éclairantes, en particulier en matière de lutte contre toutes les formes de violences. En parler, en débattre est plus que jamais nécessaire. Améliorer le cadre législatif est indispensable, car des réponses concrètes sont attendues aujourd'hui par toutes les femmes en souffrance. Ne les oublions pas

ni de « crimes passionnels ». Nous n'emploierons aucun de ces termes minimisant la réalité d'une situation insoutenable, celle de ces femmes battues à qui, un jour, leur conjoint ôte la vie. Nous ne tolérerons plus que l'espace politique ignore cette violence systémique, nourrie par un patriarcat ancestral qui laisse penser à de nombreux hommes qu'ils ont droit de vie et de mort sur leur compagne, conjointe ou ex-conjointe.

Depuis le jour où un élu régional s'en est pris au voile d'une mère musulmane accompagnatrice de sortie scolaire et la polémique qui s'est ensuivie, statistiquement,

concrète des femmes battues. Il y a urgence à agir ! Ces violences s'exercent dans tous les milieux sociaux, à tous les âges et sur l'ensemble du territoire, et elles ne semblent pas décroître.

par leur conjoint est passé de 71 en 2003 à 44 en 2019. Il y a lieu de saluer le travail de notre collègue député Aurélien Pradié et le dépôt par ses soins de la présente proposition de loi. Celle-ci dégage en effet de véritables solutions de fond pour combattre les féminicides, quand le Gouvernement paraît se contenter de faire de la communication sans effets concrets. On attend les conclusions du fameux Grenelle Nos politiques publiques ne sont tout simplement pas à la hauteur, tant sur le plan budgétaire qu'en termes d'arsenal juridique. Nous n'avons consacré cette année que 79 millions d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes, alors même que celle-ci devait être l'une des grandes causes du mandat du président Macron. Vous conviendrez, mes chers collègues, qu'il s'agit là d'une dépense résiduelle au regard du budget total de l'État. À titre de comparaison, rappelons que nos voisins espagnols, eux, mettent en oeuvre des stratégies de long terme, au travers de plans quinquennaux dotés de quelque 1 milliard d'euros. Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 500 millions d'euros par an seraient nécessaires pour protéger les femmes qui portent plainte, et 1,1 milliard d'euros pour protéger toutes les femmes en danger. Il est à espérer que l'exécutif aura ces chiffres en tête lorsque la dernière main sera mise au projet de loi de finances pour Notre arsenal juridique se révèle lui aussi insuffisant face aux dangers que tant de femmes courent au quotidien au sein même de leur foyer. cette proposition de loi vont dans le bon sens. Je pense à la réforme de l'ordonnance de protection. Actuellement, la durée moyenne de délivrance est de 42 jours. Ramener légalement le délai à 144 heures sera un gage de protection renforcée pour les victimes. En outre, le fait que ce dispositif puisse désormais être sollicité par tout moyen, sans dépôt de plainte préalable, devrait faciliter sa mise en oeuvre. L'aide personnalisée au logement pour les personnes cibles de violences conjugales ou l'extension du déploiement du téléphone grave danger sont aussi de de véritables progrès. Ajoutons que, si la répression des violences conjugales est évidemment un devoir, elle restera insuffisante si elle n'est pas accompagnée par la formation des personnels accueillant les victimes de ces violences et par l'éducation de nos enfants, dès le plus jeune âge, à l'égalité entre garçons et filles, entre hommes et femmes, pour en finir, s'il est possible, avec le fléau de la domination masculine.

Yaroslava, Taïna, Moumna, Leïla, Gulçin, Nadine et aux dizaines d'autres femmes mortes sous les coups de leur conjoint. Que nul ne les oublie !

trop longtemps, la société a tu la réalité des violences au sein de la famille. Leur persistance ne peut être ignorée et nous impose d'agir. Ce fléau n'est ni acceptable ni tolérable. Il est encore moins supportable lorsque l'on apprend que, dans un grand nombre de cas, les victimes décédées avaient signalé les violences dont elles faisaient l'objet auprès des autorités.

Les violences au sein de la famille tuent aussi les enfants : l'an dernier, 21 enfants sont ainsi décédés, tués par un de leurs parents. Ces chiffres sont connus. Ils sont terribles. Ils nous obligent. Ces chiffres sont le résultat effrayant de notre incapacité collective à protéger ces femmes- le plus souvent -, parfois ces hommes, ces enfants, victimes d'un conjoint, d'un ex-conjoint ou d'un parent violent qui se transforme peu à peu en assassin. Il ne faut pas oublier qu'à toutes ces vies ôtées s'ajoutent toutes celles qui sont brisées pour toujours : celles des victimes qui ne sont heureusement pas décédées, mais dont les cicatrices ne se refermeront jamais, celles des enfants qui ont également été victimes de violences ou qui ont enterré un de leurs parents et dont l'autre est en prison. Cette réalité insupportable doit faire l'objet d'un combat sans relâche et la République doit se montrer à la hauteur. Ce combat ne saurait être entaché de divergences partisanes : l'urgence et la gravité de la situation exigent de transcender les sensibilités politiques qui peuvent, par ailleurs, nous opposer. De même, ce combat ne peut se borner à des déclamations : il exige l'action, ici et maintenant, notamment au sein de notre assemblée. Ce n'est qu'en agissant, dans cet hémicycle, par la discussion et le vote des réponses susceptibles de diminuer le nombre des victimes de violences intrafamiliales. Tant que tous les moyens juridiques, humains et budgétaires n'auront pas été établis, notre devoir d'élus, en particulier de législateurs, ne sera pas accompli. proposition de loi, que l'Assemblée nationale a adoptée à l'unanimité le 15 octobre dernier, se compose d'un volet pénal, dont la mesure phare est la généralisation du bracelet anti-rapprochement, d'un volet civil, visant à renforcer le dispositif de l'ordonnance de protection, et d'un volet relatif au relogement des victimes de violences familiales. En ce qui concerne plus particulièrement les mesures civiles, je me réjouis que le texte tende à accélérer la délivrance de l'ordonnance de protection et à enrichir son contenu. Créée en 2010, l'ordonnance de protection permet à un juge aux affaires familiales d'ordonner, dans un bref délai, des mesures destinées à protéger une personne quand il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est la victime de violences conjugales et qu'elle court un grave danger. Ces mesures peuvent consister, par exemple, à évincer le conjoint violent du domicile conjugal ou à lui interdire d'entrer en contact avec la victime. Pour accélérer la procédure, la proposition de loi prévoit que le juge aux affaires familiales devra délivrer l'ordonnance dans un délai maximal de six jours à compter du moment où il a fixé la date de l'audience. Le texte vise également à lever les obstacles à la délivrance d'une ordonnance de protection en précisant qu'un dépôt de plainte n'est pas nécessaire et que l'ordonnance peut concerner un couple qui n'a jamais cohabité. « Toutes les violences ont un lendemain », écrivait Victor Hugo. Ce lendemain doit être apaisé et synonyme de justice pour celles qui subissent ces violences au plus profond de leur être. Ce lendemain doit être synonyme de tourments et de sanctions pour ceux qui, à travers la violence physique, ne sont que l'incarnation de la pire des lâchetés. La peur, la honte et la culpabilité doivent définitivement changer de camp. camp. Approuvant sans réserve l'objet de ce texte, les membres du groupe Les Indépendants le voteront à l'unanimité. La parole

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit ce soir concerne malheureusement toutes les couches sociales de la population, ainsi que tous les territoires. Les violences au sein de la famille- contre les femmes, dans une très large majorité des cas -touchent aussi bien les milieux modestes que des familles plus aisées, les zones urbaines que les territoires ruraux.

Pourtant, le législateur n'est pas resté inactif en la matière. En effet, la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a profondément amélioré notre droit. Comme la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, ce texte a modifié tant notre droit civil que notre droit répressif. Il a introduit d'importantes innovations, comme l'ordonnance de protection, que la présente proposition de loi tend à faire évoluer.

sur des sujets aussi graves, nous devons travailler collectivement, guidés par la volonté absolue de protéger les victimes, sans considération de nos étiquettes partisanes. Pour l'essentiel, les interventions des orateurs

mais elle nous oblige à être rigoureux, c'est-à-dire à ne voter que des dispositions effectivement normatives et, surtout, applicables concrètement. Susciter de faux espoirs chez les victimes est sans doute le principal des écueils que nous devons Notre rapporteur a parfaitement respecté ces impératifs. L'exercice n'était pourtant pas aisé. Je tiens à rendre hommage à la qualité du travail réalisé par notre collègue Marie Mercier, dont chacun connaît l'engagement sur ces sujets. Les modifications proposées en commission étaient indispensables. Elles permettent de débattre cet après-midi d'un texte bien plus abouti, juridiquement plus précis et moins « bavard

Concernant le volet civil, il est essentiellement question de l'ordonnance de protection, outil à la disposition des juges aux affaires familiales depuis la loi du 9 juillet 2010. L'ordonnance de protection est L'ordonnance de protection est une mesure très particulière. Elle est hybride : c'est une décision rendue par un juge civil, le JAF, qui évoque, par les mesures qu'elle peut contenir, une décision de nature pénale. Le JAF peut notamment ordonner des interdictions de rapprochement, contrôlées par un bracelet électronique, ainsi que des interdictions de paraître en certains lieux, comme pourrait le faire le juge répressif dans le cadre d'un contrôle judiciaire. les JAF utilisent-ils correctement et suffisamment cet outil ? Apparemment, non. D'abord, en pratique, certaines juridictions font du dépôt de plainte une condition de recevabilité de la demande d'ordonnance de protection. Ce n'est pourtant ni l'esprit ni la lettre de la loi de 2010. Ensuite, la moitié des demandes d'ordonnance de protection sont formées devant les JAF de seize juridictions, plutôt urbaines, alors que ces dernières regroupent à peine plus d'un quart des affaires familiales. Le rapport de notre collègue député Aurélien Pradié signale même que « 10 % des juridictions n'ont jamais rendu aucune décision en dix ans ». Il indique, en outre, que « la difficile montée en charge de l'ordonnance de protection » tient « toujours à un déficit de formation des juges aux affaires familiales appelés à les édicter. » C'est vrai ! Concernant le volet pénal, l'article 2 du texte complète le contenu de l'ordonnance de protection par trois mesures nouvelles, relevant plus traditionnellement du droit pénal. Le JAF pourrait notamment ordonner le port d'un bracelet anti-rapprochement, avec le consentement des deux parties. Au travers de la présente proposition de loi, nous entendons améliorer les conditions de délivrance et l'efficacité de l'ordonnance de protection.

le rôle du JAF en la matière n'est pas aisé, mais tout l'intérêt du système actuel repose sur le fait que ce juge du siège dispose d'une vision globale de la situation d'urgence et d'une palette d'outils pour protéger rapidement les victimes. Nous ne serons donc pas favorables à ces amendements. les modifications proposées de l'article 8 afin d'encourager le recours au dispositif de téléprotection communément appelé « téléphone grave danger » vont dans le bon sens. Pour que le téléphone grave danger fonctionne correctement, il doit continuer à être attribué uniquement dans les situations qui le nécessitent. Généraliser son attribution conduirait à perdre l'efficacité immédiate de l'intervention des policiers ou des gendarmes lorsqu'il est activé par la victime. Certaines des mesures que je viens d'évoquer sont appliquées chez nos voisins européens, notamment en Espagne, qui a été pionnière sur ce

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous nous félicitons que le Sénat puisse examiner aujourd'hui cette importante proposition de loi. J'espère que le débat en séance permettra d'améliorer encore

mes chers collègues, le Sénat examine aujourd'hui la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille. Dans le contexte mortifère que nous connaissons, ce texte apporte des solutions concrètes pour protéger rapidement et efficacement les conjoints victimes de violences et leurs enfants. Nous devons féliciter notre collègue député Aurélien Pradié de cette excellente initiative, récompensée par une adoption à l'unanimité à l'Assemblée nationale. De nombreuses dispositions- certaines figurent déjà dans le code civil, mais leur portée est renforcée -permettent de mettre à l'écart le conjoint violent, qu'il s'agisse de l'attribution de la jouissance du domicile familial aux victimes, de l'interdiction faite au conjoint présumé violent de se rendre dans certains lieux que la victime fréquente de façon habituelle, de la modulation du droit de visite et d'hébergement, sous dispositif électronique anti-rapprochement, qui fera toutefois l'objet d'une évaluation préalable avant son éventuelle pérennisation, ou de l'exclusion de la médiation familiale quand des violences ont été alléguées, et non plus commises. Ces mesures pragmatiques devraient démontrer toute leur pertinence dans la lutte implacable que nous menons contre les violences au sein de la famille. Elles répondent à l'objectif majeur de protéger l'intégrité physique de la femme et des enfants du couple et elles sont, à n'en pas douter, parfaitement conformes aux recommandations formulées à plusieurs reprises par la délégation aux droits des femmes du Sénat.

Si la question des violences conjugales est au centre de nos débats aujourd'hui, celle des violences subies par les enfants en est indissociable. Dans près de 70 % des cas, en effet, la violence conjugale, qu'elle prenne la forme d'agressions physiques, verbales, sexuelles ou psychologiques, se déroule devant les enfants. Dans un cas sur deux, ils la subissent directement. Cette violence peut parfois se traduire par une agression sexuelle ou un viol. Dans les cas les plus dramatiques, elle entraîne la mort de l'enfant. Notre collègue député Aurélien Pradié rapporte le chiffre de 25 décès d'enfants en 2017. De nombreuses études confirment l'impact psychotraumatique des violences conjugales sur l'enfant, cet impact variant selon le degré d'exposition à ces violences, l'âge et le sexe de l'enfant. Toutes soulignent l'altération de sa santé, de son développement affectif, physique ou cognitif et de ses conduites, l'enfant manifestant notamment des problèmes « extériorisés » d'agressivité ou d'usage de la violence ou « intériorisés », comme la dépression et la propension à être victime. Pour l'adolescent, les conséquences sont principalement des problèmes accrus de manque de confiance et d'estime de soi et le développement de comportements à risques, dont la dépendance aux psychotropes. En tout état de cause, les enfants et adolescents exposés présentent un risque élevé de reproduire les comportements violents à l'âge adulte, comme le relève l'Observatoire national de l'enfance en danger. Coconstruite avec des juristes et les acteurs associatifs, la proposition de loi d'Aurélien Pradié représente incontestablement une avancée majeure dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Toutefois, il nous faudra, j'en suis convaincue, réfléchir dans un second temps à une inflexion de certaines dispositions de notre législation, notamment en matière civile. Dans le cadre de ses travaux récents, la délégation aux droits des femmes du Sénat a, par exemple, jugé indispensable une mise en cohérence de notre législation pénale, très protectrice, avec notre législation civile, notamment le droit de la famille, qui ne prend pas suffisamment en compte les situations de violences intrafamiliales. C'est particulièrement vrai au moment de la séparation des parents, où trop souvent prévaut le modèle unique du droit de la famille, celui de la coparentalité, en vertu duquel le statut de parent est maintenu, quelles que soient les circonstances. La question de la pertinence de la résidence alternée systématique doit par ailleurs être posée. Il en est de même de la question de l'articulation de la médiation pénale, exclue en cas de violences conjugales, et de la médiation familiale, option qui demeure ouverte quand les faits de violences sont seulement allégués et non pas commis. Sur ce point, la proposition de loi Pradié apporte une réponse précise, dont nous pouvons nous féliciter. Enfin, nous devrons réfléchir à l'évolution éventuelle de l'autorité parentale, pouvant aller jusqu'au retrait total de celle-ci, car nous savons bien qu'elle peut être un moyen, pour le parent violent, de maintenir son emprise sur les membres les plus vulnérables de la famille, c'est-à-dire les enfants. À ce sujet, je rappelle que la délégation aux droits des femmes avait recommandé au garde des sceaux, dans son rapport d'information de 2016, « de diligenter une mission d'information sur le retrait total de l'autorité parentale par décision expresse du jugement pénal, à l'encontre des père ou mère qui auraient été condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent J'ajouterai pour conclure que nous ne devons pas négliger la possibilité de développer une offre de soins psychotraumatiques destinée aux enfants sur l'ensemble du territoire. L'accompagnement et le soutien psychologique des enfants sont indispensables pour les aider à se reconstruire et à comprendre les faits subis par le parent victime de violences conjugales ou par eux-mêmes, afin qu'ils ne risquent pas de devenir à leur tour des adultes maltraitants. La parole

et veille à rendre aux victimes une dignité souvent mise à mal par les titres racoleurs des médias. Madame la ministre, depuis deux mois, nous essayons de suivre le Gouvernement.

mais, madame la ministre, nous attendons de vous que vous disiez aux magistrats, à l'institution judiciaire, qu'il faut changer de pratique, changer de regard sur les femmes et enfin les croire ! Quand une femme dit qu'elle a peur, c'est qu'elle est en danger, ce n'est pas qu'elle cherche

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue député Aurélien Pradié permet de poser les premières fondations d'une politique de défense des victimes de violences conjugales. Il était temps À Bordeaux, le 21 octobre, une femme de 35 ans s'écroulait dans l'escalier de son immeuble, un couteau planté dans le coeur et des traces de violences autour du cou. Son ancien compagnon, déjà connu pour des faits de violences conjugales, est toujours activement recherché. En 2018, 121 femmes ont péri sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Nous avons déjà dépassé ce chiffre cette année : triste record, dont nous commençons à comprendre les raisons. Oui, il faut une réponse de la justice,

Il lui faut un courage inouï pour accepter de témoigner de la violence qui se déploie dans son intimité, remettre en question son univers familial. En moyenne, les femmes retirent leur plainte sept fois,

date de sa mise en service. Cela a abouti au dépôt d'une plainte dans 33 % des cas. Les victimes peuvent ainsi prendre rendez-vous avec l'enquêteur concerné et ne pas subir la salle d'attente et le délai de prise en charge. De tels dispositifs doivent être étendus. Si une femme décide de déposer plainte, c'est aussi parce qu'elle a peur pour ses enfants, dont elle ne veut pas risquer de perdre la garde. On oublie trop souvent ces victimes collatérales,

Les traces de coups ne sont pas toujours apparentes et, même si elles le sont, les enfants sont experts pour les dissimuler : il est trop difficile d'expliquer ce qui se passe à la maison. Cependant, des yeux n'oublient pas ce qu'ils ont vu, ni des oreilles ce qu'elles ont entendu, et ce quel que soit l'âge. Ce souvenir va évidemment transformer leur comportement au quotidien : les enfants victimes collatérales de violences conjugales sont quinze fois plus susceptibles que les autres d'être victimes de harcèlement ou de devenir eux-mêmes des prédateurs.

La prévention de la maltraitance est ainsi une prévention de la délinquance future. Nous devons agir vite, et nous le pouvons ! Il s'agit tout d'abord de former les enseignants et les médecins à repérer les signaux faibles, ceux que l'on peut détecter dans le quotidien d'un enfant décrocheur ou en cas de changement de comportement.

Nous devons mettre les moyens financiers à la hauteur des besoins matériels, aider la police et la gendarmerie à développer leurs programmes de sensibilisation et de prévention, qui fonctionnent déjà avec succès sur certains de nos territoires, et continuer à former à l'écoute

Au pays d'Olympe de Gouges, cette évolution préoccupante nous oblige. Aussi je me réjouis que nous examinions aujourd'hui la proposition de loi de notre collègue député Aurélien Pradié, dont je salue l'engagement et la présence dans nos tribunes.

le groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale avait déjà inscrit l'examen dans le cadre de sa niche parlementaire. Dès lors, le Gouvernement ne pouvait que réserver un accueil favorable à ce texte et, par l'enclenchement de la procédure accélérée, permettre son entrée en vigueur rapide. Il y a donc là un élan collectif, une volonté partagée et le souci d'agir avec efficacité. On ne peut que s'en réjouir. Il est vrai qu'il était urgent d'interroger l'efficacité de nos dispositifs. La proposition de loi d'Aurélien Pradié répond à cette exigence. Je pense particulièrement aux dispositions relatives aux ordonnances de protection, à la possibilité d'y recourir sans condition de dépôt préalable d'une plainte, à la réduction de leur délai de délivrance, à l'extension de leur champ.

Saluons également les dispositifs d'accès au logement pour les personnes victimes de violences conjugales. Non, la proposition de loi d'Aurélien Pradié n'est pas une petite loi toutefois vrai que, au-delà de ce texte, comme nous l'avons relevé au sein de la délégation aux droits des femmes, chère Annick Billon, la sensibilisation et la prévention des violences intrafamiliales demeurent des sujets de préoccupation sur lesquels il nous faudra travailler.

si j'en juge par l'échange que nous avons eu après le rappel au règlement de Jean-Pierre Sueur, mais il y a urgence à agir ! Voilà pourquoi, madame la ministre, je tiens à appeler votre attention sur un point essentiel

Il y va de la crédibilité de l'action publique contre un fléau qui n'a plus sa place dans notre société et qui déshonore notre République. La discussion

dès la petite enfance. Sensibiliser, éduquer, informer, former est donc incontournable en matière de prévention. Cela doit commencer à l'école, se poursuivre au collège

Lors de la journée défense et citoyenneté (JDC), les jeunes Français reçoivent un enseignement « respectueux de l'égalité entre les sexes », précise l'article L. 114-3 du code du service national. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté, aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. Au cours de cette journée, il est délivré une information générale sur le don d'organes, sur la prévention des conduites à risque pour la santé et sur la sécurité routière. Dès lors, il me semble opportun qu'une information soit également dispensée à cette occasion sur des sujets essentiels comme l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les préjugés sexistes, la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Je rappelle que plus de 1 500 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou partenaire ces dix dernières années. Cela me paraît au moins aussi important que la sensibilisation à la sécurité routière dispensée aux jeunes Français lors de cette journée. La sensibilisation aux préjugés sexistes et aux violences à l'égard des femmes fait bien partie, me semble-t-il, de l'indispensable sensibilisation aux droits et devoirs liés à la citoyenneté.

La main courante et la plainte n'ont évidemment pas les mêmes effets. C'est bien pour cela qu'elles coexistent. La main courante ne déclenche aucune action de l'autorité publique. Or, dans les situations de violences, il est important d'apporter une réponse. Je ne souhaite pas bien sûr empêcher les victimes de déposer une main courante ; elles pourront toujours le faire, cela va de soi. Je souhaite juste qu'elles ne soient pas dissuadées de porter plainte, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Cet amendement vise donc à éviter de substituer au dépôt de plainte une simple inscription dans le registre des mains courantes. Là encore, ma chère collègue, je comprends parfaitement votre préoccupation. De trop nombreuses victimes rencontrent effectivement des difficultés au moment de déposer une plainte. On leur propose alors de déposer une main courante. Cependant, l'adoption de cet amendement ne résoudrait pas la difficulté que rencontrent les femmes sur le terrain, d'abord parce que le code de procédure pénale est très clair- la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales -, ensuite parce que son interprétation risque de se révéler difficile si la victime, une fois pleinement informée des enjeux du dépôt de la plainte, souhaite finalement non plus porter plainte, mais effectuer un simple signalement des faits. Devra-t-on l'obliger à

Ce protocole, qui a été élaboré avec le ministère de l'intérieur et qui comprend quatre articles et un préambule, précise que le dépôt d'une plainte, suivie d'une enquête judiciaire, demeure le principe,

que constituent les violences au sein du couple, de sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de protéger les victimes et les enfants. Plusieurs dispositions ont également permis de s'attaquer à la source même des violences à l'égard des femmes. Je veux parler des inégalités entre les femmes et les hommes, ainsi que des stéréotypes sexistes,

car c'est dès le plus jeune âge que les stéréotypes sexistes doivent être combattus. Ils sont partout, dans la vie de tous les jours, dans les rayons de jouets, mais aussi dans les manuels scolaires, etc. À cet égard, lisez les rapports de la délégation aux droits des femmes : vous verrez où

-qu'« une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes, et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée

Et je puis attester ici que les réactions sont largement positives et qu'elles incitent à l'optimisme. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que ces informations

2006. J'en viens à la loi de juillet 2010. L'ordonnance de protection constituait, dans notre esprit, une réelle évolution de notre droit, qui se dotait ainsi d'un outil de protection complet et rapide

c'est-à-dire en urgence et en priorité- ce n'était peut-être pas très réaliste -et qu'elle puisse être obtenue indépendamment du dépôt de plainte- la loi est d'ailleurs claire sur ce dernier point -, mais certains magistrats, il est vrai, ont pris de mauvaises habitudes. Il était donc opportun de rappeler à l'article 1 l'état du droit sur ce point. Par ailleurs, et j'anticipe sur l'article 2, encadrer la procédure dans un délai de 144 heures, à compter de la date de la fixation de l'audience, devrait permettre au magistrat d'apprécier la recevabilité de la requête, avant que la partie défenderesse ne prenne connaissance de la démarche, ce qui devrait éviter certaines représailles. Il y a un mieux dans cette évolution, à condition que l'audience ne soit pas fixée plusieurs dizaines de jours après. Je m'interroge donc : comment faire mieux pour répondre à l'urgence, tout en respectant le contradictoire ? La parole est à Mme Marie-Pierre Monier,

Ce fléau est insupportable, d'autant plus que, dans un grand nombre de cas, la victime avait signalé les violences dont elle faisait l'objet auprès des autorités. Si des outils juridiques existent aujourd'hui, ils sont souvent mal utilisés. Il faut aller plus loin, en protégeant mieux les victimes et en renforçant les garanties matérielles et juridiques dont elles bénéficient. Le parcours des victimes est trop long. Surtout, il est bien souvent jonché d'obstacles : refus de plainte, remise en question de la gravité des faits, culpabilisation des victimes, moqueries. Ce n'est plus acceptable. J'en profite pour saluer l'immense courage d'Adèle Haenel, qui vient de porter un nouveau coup historique à l'insupportable loi du silence qu'il nous faut briser. Désormais, j'en suis certaine, plus rien ne sera comme avant. Je veux rendre hommage à sa justesse bouleversante. Au-delà de l'occasion de libérer la parole qu'elle nous offre, elle nous rappelle que le combat contre les violences faites aux femmes ne se gagnera que si nous parvenons à déconstruire les stéréotypes de genre, car ce sont bien eux qui inscrivent en chacun de nous, dès l'enfance, la possibilité de ces violences. Pour les combattre, nous devons irriguer toutes les politiques publiques. C'est pourquoi un vaste projet de loi sur le sujet, associant police, gendarmerie, justice, services sociaux, collectivités locales, services de santé, éducation nationale associations militantes aurait été plus fort. Malgré tout, il convient de soutenir les dispositions proposées, car elles vont dans le bon sens, mais il faudra prévoir les moyens que requiert la mise en oeuvre de cette proposition de loi lors de l'examen du projet de loi de finances. des moyens pour faire fonctionner les associations de terrain, qui maillent le territoire et jouent un rôle majeur d'accompagnement ; des moyens pour la formation des policiers et des gendarmes, qui sont en première ligne pour accueillir les femmes victimes de violences, car ils ont besoin de soutien pour jouer leur rôle de service public de proximité. Sans moyens supplémentaires, sans personnels formés, ce que nous votons ici ne pourra pas avoir de réel impact sur le cours des choses. La parole est à M. François Bonhomme,

En fixant à six jours le délai maximal de délivrance d'une ordonnance sans dépôt de plainte, l'ordonnance doit constituer un moyen nouveau et décisif. Or il y a encore trop de manquements graves, puisque, dans un cas sur cinq, le juge ne statue pas sur la restriction du droit d'hébergement des enfants, et, dans un cas sur deux, il ne traite pas de la question pourtant essentielle du logement. La situation actuelle n'est donc pas acceptable en l'état. Renforcer l'ordonnance de protection, c'est aussi créer une interdiction de paraître pour les auteurs de violences. Il faut les empêcher d'attendre devant l'habitation. Désormais, certains lieux entiers leur seront interdits, au-delà même du seul contact physique.

La pose d'un BAR dès l'ordonnance de protection dans un cadre préventif et pour les situations les plus graves, ainsi que la possibilité donnée au juge aux affaires familiales de décider d'agir dans un délai réduit réduit peuvent constituer une mesure déterminante pour éviter ces drames trop souvent répétés. Raccourcir les délais de prononcé des ordonnances de protection est une nécessité, tout en veillant à l'articuler avec le respect du principe du contradictoire et en rappelant la nature spécifique de la procédure civile, qui repose sur des principes différents de la procédure pénale.

Je crois, madame la garde des sceaux, que nous pouvons faire converger de manière décisive une prise de conscience très forte de ce fléau et l'impératif de lui donner une portée opérationnelle déterminante. Il est réjouissant que cette proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié soit l'occasion de faire converger nos forces, y compris et peut-être surtout quand un texte ne vient ni du Gouvernement ni de la majorité. C'est l'honneur du groupe parlementaire d'opposition à l'Assemblée nationale de nous permettre de dépasser nos différences pour réduire ce sinistre bilan de 119 femmes ayant à ce jour perdu la vie en 2019 sous les coups de leur conjoint. La parole est à M. Marc Laménie,

Cette habilitation nécessiterait évidemment au préalable le consentement de la requérante. L'obtention de l'ordonnance de protection est administrativement lourde. Une fois mise en sécurité, la victime souhaitant recourir à un tel procédé doit au préalable comprendre comment rédiger, puis soumettre une telle demande, alors même qu'elle se trouve souvent en situation de détresse et n'a pas forcément les connaissances juridiques nécessaires pour mener à bien cette mission. Afin de multiplier les chances d'obtention, il peut être pertinent que, à la demande de la victime, les associations agréées puissent formuler la demande d'ordonnance de protection. Elles sont en effet plus aguerries et mieux armées juridiquement, ayant développé une expertise procédurale en la matière. Leur rôle d'accompagnement est donc primordial, particulièrement dans des situations d'urgence. Les associations agréées accomplissent un travail formidable dans les territoires. Elles apportent non seulement une aide juridique aux victimes, mais également un soutien psychologique indispensable.

efficace. Quel est l'avis de la commission ? avec l'accord de la victime, la constitue partie demanderesse pour une ordonnance qui devrait en principe bénéficier à une autre personne, et qui ne serait paradoxalement pas partie à la procédure. En outre, en l'état actuel de la rédaction du texte, une telle éventualité est incompatible avec le dispositif retenu qui vise systématiquement la partie demanderesse comme unique bénéficiaire. L'association serait bénéficiaire de l'ordonnance de protection, et non plus la victime. C'est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable

Mme le rapporteur. Il n'y a pas de mandat qui soit donné à l'association par la victime. L'association ne peut faire la démarche pour la victime, puisque l'ordonnance de protection sera rendue au nom de cette dernière. Ce n'est pas comme avec un avocat.

madame la ministre,

donc de distinguer la représentation, dont le monopole appartient aux avocats, et l'accompagnement, qui peut parfaitement être exercé par les associations.

à pouvoir la demander. ; il permet à la victime, d'une part d'être accompagnée, d'autre part d'être représentée par l'avocat. C'est largement suffisant pour porter la défense des personnes concernées.

L'une d'elles, très ambitieuse, est de réduire à six jours le délai au-delà duquel le juge aux affaires familiales doit rendre sa décision sur l'ordonnance de protection, celle-ci statuant

efficace. Quel est l'avis de la commission ?

mais requiert des évolutions en matière d'aide juridictionnelle, afin que celle-ci soit accordée dès la demande de l'ordonnance de protection et non plus au moment de sa délivrance. Pour cette question de faisabilité, nous demandons l'avis du Gouvernement.

La voie administrative mérite donc d'être creusée comme l'un des moyens de saisir très rapidement, dans un débat contradictoire, les deux parties, pour que la décision puisse être rendue sans délai et de manière efficace.

En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 27 voix pour, aucune voix contre -à la nomination de M. Yves Le Breton aux fonctions de directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.